L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret,

anniversaire, tous les jeunes reçoivent une convocation pour participer à la JDC et ainsi s'informer des droits des citoyens, de leurs devoirs et du fonctionnement des institutions. Le ministère des affaires étrangères a décidé il y a quelques années, pour des raisons budgétaires, de supprimer les JDC tout en autorisant leur maintien dans les pays où le chef de poste diplomatique et consulaire le jugerait utile et possible. L'année dernière, en raison de la pandémie, la JDC a été supprimée pour tous les jeunes Français de l'étranger, y compris dans les pays où l'ambassade avait décidé de la maintenir, tandis qu'elle se tenait en ligne pour les jeunes résidant en France. diplomatiques et consulaires ont délivré une attestation provisoire de report permettant aux jeunes Français résidant à l'étranger de justifier de la régularité de leur situation au regard de la loi et ainsi de s'inscrire aux concours et examens, et de passer leur permis de conduire. ailleurs appris en avril dernier que le ministère des armées et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères travailleraient à une adaptation du dispositif de JDC en ligne à l'attention des jeunes Français établis hors de France. je souhaiterais donc savoir si les modifications techniques et réglementaires nécessaires ont été adoptées : le système est-il en place ? Si tel n'est pas le cas, comment la JDC est-elle organisée cette année pour les jeunes Français de l'étranger, en particulier dans les pays où la situation sanitaire est encore fortement dégradée ? La parole

de délitement du lien social et un individualisme croissant ; la JDC fait partie, à mon sens, des remèdes qui doivent être absolument préservés. On ne peut pas à la fois verser des larmes de crocodile sur

là où les plus grosses communautés françaises sont présentes, que ce soit à Londres, à Bruxelles, ou encore à Genève. C'est important de pouvoir le faire : comptez sur moi pour le redire avec insistance à nos postes

propositions ont été émises dans le débat public ; je les reprends bien volontiers à mon compte. De la même façon, il est essentiel qu'un jeune Français établi hors de France ait les mêmes droits qu'un jeune établi en France. Madame la sénatrice, nous allons poursuivre dans cette voie

Madame la secrétaire d'État, êtes-vous consciente et soucieuse de ce qui se passe dans nos villages ? Des classes ou des écoles continuent de fermer sans qu'aucune consultation n'ait été engagée avec les maires. Cela suscite l'émoi et l'incompréhension des familles, ainsi qu'une rupture de confiance entre les élus et le Gouvernement que vous représentez. Il y a tout juste un an, le Gouvernement avait pourtant annoncé qu'en raison des circonstances sanitaires exceptionnelles il n'y aurait aucune fermeture de classe en milieu rural à l'école primaire sans l'accord préalable du maire. Les hussards de la République, dans les Vosges comme sur tout le territoire national, ne ménagent pas leur peine au quotidien pour contribuer au maintien d'un enseignement de qualité, pour promouvoir l'égalité des chances et l'attractivité de nos communes. Les décisions de suppression de classes ou d'écoles portent préjudice à ces objectifs et suscitent de nombreuses difficultés d'ordre juridique, organisationnel et budgétaire.

On ne rouvre jamais une classe, une école, avec la même promptitude qu'on ne la ferme, tant les obstacles administratifs, budgétaires et parfois politiques sont nombreux. Madame la secrétaire d'État, ne convient-il pas d'envisager un moratoire des fermetures de classes ou d'écoles ? À défaut, quelles mesures de compensation et d'accompagnement pourriez-vous proposer aux maires afin de pallier les conséquences, notamment financières, de vos décisions unilatérales ?

C'est la raison pour laquelle, depuis le début de ce quinquennat, nous n'avons jamais cessé d'augmenter les moyens consacrés au premier degré, et ce dans un contexte de forte baisse démographique

aucune fermeture d'école en milieu rural ne peut intervenir sans l'accord du maire. C'était le cas et cela reste le cas ! L'engagement de ne fermer aucune classe en milieu rural

Depuis lors, la situation s'est aggravée : à certains endroits, la navigabilité de la Rance s'est détériorée, ce qui porte préjudice aux riverains et aux communes, ainsi qu'à leur attractivité touristique. En matière d'atteintes à la biodiversité et au patrimoine naturel, le constat suscite des interrogations. Je le redis donc aujourd'hui : il y a urgence Pour y répondre, une voie complémentaire au plan de désenvasement peut être explorée. En effet, depuis 2019, la Commission européenne se montre favorable à la revalorisation au tarif « énergie renouvelable » de l'électricité produite par l'usine marémotrice de la Rance (UMR), site unique en Europe. Si la levée de ce blocage a été accueillie avec enthousiasme par l'ensemble des parties prenantes, le ministère de l'environnement a néanmoins précisé que « la création d'une fiscalité écologique spécifique sur l'électricité produite par l'usine marémotrice de la Rance n'est pas l'option à privilégier à court terme », préférant renvoyer au plan de gestion des sédiments. Pourtant, depuis le 1 juillet dernier, l'article L. 211-2 du code de l'énergie dispose clairement que l'énergie marémotrice est une énergie renouvelable. Par ailleurs, EDF, concessionnaire de l'UMR, a réitéré son attachement à cet équipement Pour autant, on sait que le projet de réorganisation du groupe, dit « Hercule », qui est actuellement suspendu, pourrait affecter le passage en tarification verte de l'énergie produite. L'UMR pourrait ainsi être classée parmi les barrages hydroélectriques, plutôt qu'au sein de la branche « énergies renouvelables », ce qui constituerait un nouveau frein pour la valorisation de l'énergie produite par l'UMR et compliquerait ainsi les investissements à réaliser. C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, je souhaite connaître votre position sur ce sujet : allez-vous soutenir la tarification verte pour l'électricité produite par l'UMR, en cohérence avec les dispositions du code de l'énergie ? La parole

du contrat de concession. Or le droit des concessions n'autorise pas à modifier substantiellement l'économie d'un contrat en cours, à moins d'une nouvelle mise en concurrence. Par ailleurs, il n'apparaît sans doute pas judicieux de mettre en place un tel soutien public pour une concession hydroélectrique alors que la France fait face à à deux mises en demeure de la Commission européenne. Enfin, la classification en concession hydroélectrique et la qualification d'énergie renouvelable sont absolument indépendantes d'une éventuelle réorganisation du groupe EDF. Madame la sénatrice, il convient donc, à ce stade, de poursuivre et de soutenir les travaux en cours pour que des solutions pérennes de lutte contre l'envasement de l'estuaire soient identifiées

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur les moyens de l'Office français de la biodiversité (OFB) dans les Alpes-Maritimes. Alors que les services de l'OFB dans ce département devraient compter 17 inspecteurs de l'environnement, on y dénombre seulement 8 fonctionnaires à temps plein et 1 à mi-temps. La police de l'environnement et la surveillance de la biodiversité sont ainsi assurées ainsi assurées par des inspecteurs en sous-effectif. Cela rend leurs missions particulièrement difficiles à accomplir, d'autant qu'ils couvrent les milieux aquatiques, terrestres et maritimes. L'une de ces difficultés s'exprime tout particulièrement lorsqu'un inspecteur de l'environnement doit se rendre auprès d'un éleveur après une attaque de loup afin de réaliser le constat de dommages. Si les inspecteurs sont naturellement qualifiés pour ces missions, elles ont par le passé été confiées à des ouvriers forestiers formés par les inspecteurs de l'environnement de l'ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage, ce qui permettait aux inspecteurs de se concentrer sur leur coeur de métier. En demi-effectif, les agents de l'OFB ne sont pas assez nombreux pour réaliser l'ensemble des constats, alors même que la prédation est particulièrement intense tout au long de l'année dans les Alpes-Maritimes. Ces allers-retours, qui requièrent plusieurs heures de marche vers les zones d'estive ou de pâturage, les limitent dans leurs missions.

d'État, entendez-vous modifier la méthode de déclaration afin de passer à un téléconstat, dispositif défendu tant par les éleveurs, qui n'ont pas tous de matériel numérique, que par les inspecteurs de l'environnement, capables de réaliser le diagnostic de l'attaque par téléphone sans avoir à se déplacer dans des zones de montagne très reculées

Dans cette optique, un dispositif de constat déclaratif des dégâts a été expérimenté dans certaines zones et pourrait être étendu. Nous étudions par ailleurs avec le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

projet de loi de finances pour 2022, puisque j'ai eu la joie d'annoncer que les opérateurs de la biodiversité ne connaîtraient pas de réduction de schéma d'emploi cette année. Nous maintenons les effectifs, nous renforçons les moyens de manière structurelle dans le projet de loi de finances- j'en remercie les parlementaires -et

Mme Dominique Estrosi Sassone, pour la réplique. Madame la secrétaire d'État, vous dites que vous maintenez les emplois, mais vous ne les augmentez pas ! Je viens de vous faire la démonstration que, dans les Alpes-Maritimes, les fonctionnaires qui travaillent pour l'Office français de la biodiversité sont nettement en sous-effectif : de fait,

De plus en plus de nos concitoyens, dans mon département, mais aussi ailleurs, se sont manifestés depuis que ma question a été publiée : cela montre que ces retards sont importants. Des gens modestes, voire très modestes, veulent changer leur chaudière ou isoler leur logement ; ils ont engagé des travaux après approbation de leur dossier par l'ANAH, mais les remboursements ne viennent pas

très concrète, comment vous comptez améliorer le traitement de ces dossiers et permettre un paiement extrêmement rapide une fois les travaux réalisés et les factures éditées. La parole

En effet, s'il relève du domaine public de la ville, il assure depuis 1973 un rôle de premier plan dans la mobilité et l'attractivité économique de toute la métropole.

installer des carrefours avec des feux tricolores, des passages piétons, des pistes cyclables, des espaces verts, voire des commerces- tout cela, sur le périphérique parisien D'après une étude réalisée par la ville à l'automne 2020, rendue publique au mois de janvier 2021, les usagers du boulevard périphérique, qui ne sont bien entendu pas tous parisiens, sont très majoritairement hostiles à ces éventuelles modifications. Compte tenu de l'évolution et de l'importance de cette voie de circulation, compte tenu aussi de son impact, qui dépasse la population installée à l'intérieur de cet anneau routier, je tiens à interroger le Gouvernement sur l'opportunité d'engager une réflexion sur une autorité partagée de cette ceinture périphérique, qui reste la plus empruntée d'Europe.

ailleurs, le boulevard périphérique étant un axe essentiel à la sécurité de Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, l'État peut émettre des prescriptions qui visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules, notamment de sécurité et de secours. La gouvernance de cet axe, à vocation à la fois locale et nationale, est donc claire et l'État est tout à fait vigilant au maintien de son bon fonctionnement. À ce jour, le préfet de police n'a été destinataire d'aucun dossier d'aménagement spécifique, sauf pour ce qui relève

C'est pour cette raison que le préfet de la région d'Île-de-France a mis en place une conférence stratégique sur les mobilités routières, rassemblant État et collectivités, pour constituer un véritable lieu naturel d'échanges sur ces sujets. Plusieurs initiatives et alternatives à la congestion existent dans le même temps : incitation au covoiturage, développement des transports en commun en connexion entre Paris et la banlieue, etc. L'État est pleinement mobilisé, vous le savez, puisque ce sont notamment près de 670 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour finaliser 100 % des projets de transports collectifs du contrat de plan qui seront déployés. Je précise par ailleurs, car cela a animé le débat public dernièrement, que la région peut, dans le cadre de cette conférence, faire part de ses souhaits et de ses attentes. Nous appelons donc à des échanges sereins entre collectivités et au sein des instances de dialogue existantes. La parole

ministre de la transition écologique. Depuis quelques années maintenant, les dérèglements climatiques s'accumulent sur notre territoire, comme dans le monde. À l'échelle locale, celle de mon département du Pas-de-Calais, les épisodes de sécheresse succèdent aux pluies diluviennes, qui lessivent les sols et provoquent des mouvements de terrain, des coulées de boue et des destructions matérielles importantes. Les zones rurales sont particulièrement touchées, mais souvent ignorées. Je pense ainsi à la vallée de la Canche, où une dizaine de communes ont encore été touchées au printemps En effet, si l'extension urbaine, qui implique l'artificialisation des sols, est l'une des causes premières des inondations et des coulées de boue, ce n'est pas le cas de nos campagnes. En ruralité, c'est davantage le défaut de pilotage et le manque de moyens dévolus à l'aménagement du territoire et à la concertation qui posent problème. En effet, quand les exploitants agricoles sont majoritairement en fermage, c'est-à-dire ne sont pas propriétaires des terres qu'ils exploitent, qui doit intervenir pour rétablir les obstacles empêchant le lessivage des sols ? De même, l'angle d'attaque choisi par le Gouvernement de créer des lignes budgétaires dans le plan de relance pour les propriétaires fonciers est une bonne idée. Toutefois, cela retire aux élus locaux la maîtrise de l'aménagement du territoire. Les maires, Les maires, qui ont une vue d'ensemble de l'aménagement du territoire, ne sont pas consultés et n'ont pas de pouvoir pour mener des travaux d'entretien des fossés et des noues, et replanter des haies sur les terrains privés. De nombreux acteurs travaillent isolément sur ces questions, ce qui rend inefficace la prévention des inondations. Plus problématique encore, l'absence de concertation induit des incompréhensions entre les exploitants, les pouvoirs publics et la collectivité. On a donc, d'un côté, des techniciens performants, mais non coordonnés, et, de l'autre, des élus volontaires, mais dépourvus de moyens, et des exploitants dont le rôle n'est pas la gestion des bassins versants. Pour mettre en oeuvre une politique efficace de prévention des inondations, il faut un chef d'orchestre. Les maires sont des candidats tout désignés pour ce rôle, mais le transfert de compétences en matière d'urbanisme aux établissements publics

vous m'interrogez sur les outils disponibles pour lutter avec toutes les parties prenantes contre les inondations, en particulier celles qui sont causées par les ruissellements provenant de parcelles cultivées.

pour mettre en place une stratégie globale de gestion du risque, y compris du risque inondation exceptionnelle par ruissellement, et bénéficier ainsi d'un cofinancement du fonds Barnier. Nous avons également souhaité accroître les moyens de la prévention des inondations pour soutenir encore plus les collectivités dans cette résilience des territoires.

Le soutien financier de l'État aux porteurs de projets pour l'animation des PAPI a été revalorisé. Par ailleurs, la labellisation a été simplifiée. En outre, dans le cadre de la compétence Gemapi, les collectivités peuvent engager toute action qu'elles jugent nécessaire afin de prévenir les inondations, y compris celles qui sont causées par ruissellement. Ces actions peuvent être financées à travers la taxe Gemapi. À l'échelon national, des travaux sont en cours dans le cadre de la commission mixte inondation afin de faciliter la prise en compte de l'activité agricole et des espaces naturels dans la gestion des risques d'inondation. Dans les Hauts-de-France, nos services sont pleinement mobilisés sur ces actions concrètes, qui doivent nous permettre de mieux connaître les origines et les phénomènes de ruissellement. En outre, un effort sera engagé pour mieux informer sur les différents dispositifs financiers mobilisables- fonds Barnier, fonds européens, fonds des agences de l'eau, mesures soutenues par la

Créées par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les ALEC accompagnent quotidiennement les collectivités et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'énergie et au climat dans leur champ de compétences, notamment les transports, l'urbanisme et le logement.

en les connectant davantage aux services déconcentrés de l'État et en énumérant certaines des missions qui peuvent leur être confiées. Il s'agit là d'une première avancée attendue. Cependant, il convient désormais de sécuriser fiscalement ces structures. La situation actuelle entraîne des aberrations, comme le fait que les collectivités doivent payer la TVA sur les subventions qu'elles versent à ces organismes. D'autres agences sont menacées par des redressements fiscaux. Ainsi, pour une approche globale et complète, un rescrit fiscal permettrait de lever les derniers doutes sur le régime applicable aux missions des ALEC. Un tel document permettrait de garantir la vocation première des ALEC, qui est de développer des projets sur les territoires pour susciter la demande et faire progresser l'offre, et non de se substituer au secteur concurrentiel. Madame la secrétaire

Elles contribuent à l'élaboration des documents en matière d'énergie et de climat. Elles facilitent également la mise en oeuvre des politiques locales en fournissant des indicateurs chiffrés sur les consommations et les productions énergétiques, sur les émissions de gaz à effet de serre, afin d'assurer un suivi de la mise en oeuvre de ces politiques.

intercommunale à fiscalité propre peuvent s'appuyer sur les ALEC pour mettre en avant le service public de la performance énergétique de l'habitat. Je note d'ailleurs que, dans un communiqué du 22 juillet dernier, la Flame a salué l'adoption de ces dispositions. Nous allons donc

TVA. Les ALEC peuvent tout à fait être constituées sous une forme associative et, le cas échéant, bénéficier d'exonérations applicables aux organismes sans but lucratif. L'application de ces règles ne peut cependant s'apprécier qu'au cas par cas, notamment dans le cadre de la démarche de rescrit fiscal en fonction des activités de l'ALEC, des modalités de son financement et des circonstances dans lesquelles elle intervient localement. Les services du ministère de la transition écologique et du ministère de l'économie, des finances et de la relance restent à disposition des ALEC auprès de leur fédération

Monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dans cet hémicycle sur la guerre urbaine sur fond de trafic de drogue qui se déroule dans ma ville de Cavaillon. C'était le 21 juillet dernier. Depuis, chaque jour, on déplore des tirs, des rafales de kalachnikov, des blessés qui tombent sous le coup des balles. Au regard de la gravité de la situation et de l'impérieuse nécessité d'agir fort et vite, c'est toute la chaîne police-justice qu'il est nécessaire de conforter. Les quatre cabinets d'instruction, Avignon étant pôle criminel, sont au bord de l'implosion : le tribunal correctionnel explose du fait des procédures tentaculaires de trafic de stupéfiants, alors que la cour d'assises, entre session ordinaire et sessions supplémentaires, siège de façon quasi permanente. Le procureur de la République fait ce qu'il peut, mais il manque de moyens. Manifestement, la justice est sous-dotée à Avignon. Monsieur le garde on ne lutte pas contre des trafics de cette dimension avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur. Je profite de cette occasion pour saluer le travail accompli par ces cabinets d'instruction aux côtés des services d'enquête compétents et dévoués à lutter avec acharnement contre ce fléau, qui pénalise au premier chef les habitants majoritairement paisibles de ces quartiers gangrenés. Toutefois, l'épuisement moral gagne, y compris les magistrats. Monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, il faut beaucoup plus de moyens pour la justice à Avignon, sur le temps long et sur l'ensemble de la chaîne pénale. Cela signifie plus d'effectifs, plus de personnels. Il faut des juges d'instruction, des juges correctionnels, des greffiers et des agents qui sont en capacité de traiter ces affaires qui arrivent sans cesse. Cela signifie concrètement pour Avignon la mise en place d'un cinquième pôle instructeur, la nomination de deux magistrats au tribunal correctionnel et d'un magistrat au pôle criminel. Monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre, avec le ministre de l'intérieur, vous avez déclaré vouloir faire cette guerre totale à la drogue. Encore faut-il que le Gouvernement mette les moyens pour agir fort et vite, principalement dans mon département, au tribunal de grande instance d'Avignon. La parole

à entamer la discussion du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, je me suis particulièrement intéressée au titre III de ce texte et au travail pénitentiaire. Après l'adoption du projet de loi, nombre de mesures, contenues notamment dans les articles 11 à 14, seront prises par décret et par ordonnance.

qui permet à 80 % de la population carcérale d'être éligible au travail dans le cadre d'ateliers d'excellente qualité offrant aux détenus formation, accompagnement et préparation à la sortie. Les ordonnances seront à écrire de façon collégiale.

et je ne ménage pas mes efforts pour que le travail revienne en prison. C'est bon pour le patron, c'est bon pour le détenu, c'est bon pour toute la société.

que Muret, qui est un établissement pénitentiaire que nous connaissons bien, vous et moi, sera retenu pour cette expérimentation, qui a pour but- redisons-le, car c'est un sujet qui nous est commun -d'éviter au maximum la récidive et de favoriser au mieux la réinsertion.

En effet, les juges consulaires bénévoles qui les composent alertent très souvent sur l'insuffisance des moyens de fonctionnement qui leur sont alloués. Ainsi, en 2016, le président du tribunal de commerce de Paris déplorait-il un budget de fonctionnement de 12 000 euros par an.

en période de crise sanitaire. Je pense à l'absence de bande passante suffisante pour pratiquer des visioconférences ou d'un système fiable de signature électronique : autant d'entraves qui pourraient se révéler néfastes, notamment si le nombre de faillites d'entreprises venait à augmenter, ce qui n'est pas le cas en ce moment. La justice consulaire est bénévole, ce à quoi les juges sont particulièrement attachés. Il y a cependant une différence entre exercer ses fonctions sans être rémunéré et devoir parfois payer de ses propres deniers des dépenses de fonctionnement de la structure ou encore supporter les frais afférant à sa fonction, ce qui est malheureusement fréquemment le cas. Des calculs réalisés par certains représentants des tribunaux de commerce démontrent qu'un effort budgétaire national de 1 million d'euros, soit 0,16 % du montant de l'augmentation du budget de la justice en 2020, devrait raisonnablement suffire à régler les questions financières du quotidien. à l'heure de la présentation du projet de loi de finances pour 2022, votre ministère se voit attribuer une augmentation de 8 %, ce dont je me satisfais. Pouvez-vous m'indiquer quel montant sera alloué aux juridictions commerciales ?

Souvent, quand on compare la justice- c'est un jeu que l'on aime dans notre pays -, on compare la justice allemande et la justice française. La justice française compte des juges bénévoles tribunaux de commerce, vous l'avez rappelé, mais aussi dans les juridictions prud'homales. J'en viens à la question précise que vous me posez. Le renforcement du budget, inédit depuis ans, s'est traduit par une hausse de la dotation de fonctionnement des cours d'appel et l'allocation de fonctionnement courant répartie en début de gestion a augmenté de plus de 3 % par rapport à 2020.

de commerce de Nantes, soutenues à la mi-septembre de l'année en cours, représentent 0,33 million d'euros, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année 2020. Le budget 2022 devrait permettre de garantir le niveau de soutien apporté au tribunal de commerce nantais. Pour être tout à fait complet, monsieur le sénateur, j'ajoute que le Conseil national des tribunaux de commerce travaille actuellement à l'élaboration d'un guide budgétaire, qui permettra aux présidents des tribunaux de mieux connaître la procédure d'octroi de leur budget de fonctionnement.

Ce texte offre en effet la possibilité aux communes d'être dispensées de l'élaboration d'un double des registres, à condition toutefois de justifier de conditions de sécurité renforcées nécessaires à la bonne tenue et à la sécurisation des données de l'état civil. Les conditions de sécurité des données de l'état civil et celles permettant aux mairies d'être dispensées d'établir un registre en double exemplaire ont été fixées par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 2017 relatif à l'état civil, pris après avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes. Toutefois, dans sa réponse à la question écrite n° 01643 publiée dans le du Sénat du 19 octobre 2017, la Chancellerie précise qu'un « arrêté fixant les conditions techniques de sécurité des traitements automatisés utilisés par les communes [serait] soumis à la Commission nationale de l'informatique

garde des sceaux, je vous demande de bien vouloir m'indiquer si la suppression de la tenue du second registre papier de l'état civil est bien applicable en l'état ou si, le cas échéant, vous entendez publier le texte réglementaire manquant.

qui a ouvert aux communes la faculté d'être dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des registres d'état civil. Cette possibilité a toutefois été soumise à la condition que les communes en question disposent d'un traitement automatisé de données d'état civil qui satisfont à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret. Le décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil est depuis venu préciser cette disposition, en renvoyant toutefois à un arrêté pour spécifier les modalités de mise en oeuvre précises des conditions techniques supplémentaires exigées. Les travaux préparatoires à la rédaction de cet arrêté sont en cours.

évidemment à l'objectif de cette réforme, à savoir alléger les exigences formelles qui pèsent sur les communes et leurs maires, il est indispensable que l'État s'assure que les conditions en termes de sécurité de cet allégement soient réunies. soient réunies. Pour répondre parfaitement et complètement à votre question, monsieur le sénateur, je tiens à vous assurer que cet arrêté devrait être publié dans un délai d'un an, après un travail très important de mes services auprès des mairies et des éditeurs de logiciels d'état civil.

En raison de la pandémie, les radios locales indépendantes et associatives se retrouvent dans une situation financière délicate, bien qu'elles aient bénéficié de deux aides importantes : le fonds d'aide à la diffusion hertzienne et le crédit d'impôt temporaire de 15 % en faveur des diffuseurs. Ces radios ont tout fait pour poursuivre leur travail afin d'assurer leur mission d'information et de maintenir du lien social au coeur des territoires. C'est pour cette raison qu'elles n'ont pas souhaité mettre leur personnel en chômage partiel. Leur budget repose en grande partie sur des recettes publicitaires, qui ont fondu durant la crise sanitaire. Parallèlement, leurs charges sont restées les mêmes, voire ont augmenté en raison des nouvelles contraintes techniques liées aux règles sanitaires. Certaines de ces radios locales sont actuellement dans l'attente du versement du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER), qui accuse un retard important en 2021. En effet, au lieu d'être en partie versé à la fin du printemps, il ne le sera vraisemblablement qu'en décembre prochain, après que la commission compétente se sera réunie en novembre. De plus, pour soutenir le déploiement en France du DAB+ (, ou radiodiffusion numérique), qui va nécessiter plusieurs millions d'euros d'investissements, les radios locales sollicitent la création d'une nouvelle aide, sans laquelle elles ne pourront pas en supporter le coût. Pour toutes ces raisons, il est à craindre que ces radios disparaissent, malgré les prestations de qualité qu'elles peuvent offrir. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer quelles mesures vous entendez prendre afin de continuer à les accompagner dans cette période critique, pour préserver un paysage radiophonique dense et pluraliste La parole

Mouiller, les médias locaux, à l'image des radios locales, ont joué un rôle de premier plan durant la crise sanitaire, en assurant l'information et l'accès à la culture de tous les citoyens. Les radios commerciales locales, dont les ressources publicitaires ont fortement baissé au printemps 2020, ont maintenu leur activité. Le ministère de la culture- comme vous l'avez rappelé, ce dont je vous remercie -les a accompagnées à travers deux dispositifs exceptionnels le fonds de soutien à la diffusion hertzienne, dont Collines FM a bénéficié, et le crédit d'impôt au profit des diffuseurs audiovisuels pour leurs dépenses dans la création. Les radios associatives n'ont pas été épargnées par la crise, bien que leur économie soit largement indépendante des aléas du marché publicitaire.

Les mesures d'adaptation des modalités de détermination des subventions ont été saluées par les organisations représentatives de ces radios, que j'ai d'ailleurs reçues récemment. Aucune anomalie n'a été relevée s'agissant du calendrier de versement des aides, dont bénéficient notamment la radio D4B, Radio Gâtine et Radio Val d'Or. Dans un Dans un contexte de poursuite du développement du DAB+, j'ai obtenu dans le projet de loi de finances pour 2022 une nouvelle augmentation des crédits du FSER, qui atteindront ainsi un niveau historique à 33,1 millions d'euros, soit une hausse de 1,1 million d'euros, c'est-à-dire de 3,5 %, par rapport à 2021. Je vous signale par ailleurs que les chiffres publiés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) au mois de juillet, pour le premier semestre de l'année 2021 révèlent que le marché publicitaire national des radios a retrouvé un niveau similaire à celui observé avant la crise, profite également aux radios locales, lesquelles tirent en moyenne la moitié de leur chiffre d'affaires publicitaire de ces recettes. Les dernières données relatives au marché publicitaire font également apparaître une dynamique positive pour le second semestre. Dans ce contexte, il ne me paraît pas justifié de reconduire ces dispositifs exceptionnels, conçus pour répondre à la baisse sans précédent des investissements publicitaires. Le maintien des mesures d'adaptation du FSER sera quant à lui étudié en fin d'année,

et la pandémie ont en effet entraîné d'importants bouleversements dans les habitudes de lecture des Français mais aussi dans le monde de l'édition. Cette activité culturelle, qui génère un chiffre d'affaires assez important, est toujours autant plébiscitée par nos concitoyens. Or, avec l'arrivée du numérique, le marché du livre est en pleine mutation, avec près de 400 000 titres disponibles à la vente et accessibles un ordinateur fixe, une liseuse, un smartphone, une tablette ou encore un ordinateur portable. Surtout, ce marché, en augmentation constante, a connu une hausse particulièrement notable au plus fort de l'épidémie de covid-19. Durant cette période, les chiffres communiqués par les plateformes de vente spécialisées témoignent même d'une hausse spectaculaire des achats de livres numériques, avec un nombre de téléchargements et de ventes multiplié par sept, tandis que le nombre d'commandés a été multiplié par Quant à la lecture directe sur un ordinateur, elle a triplé en volume, ce qui représente plus de 800 000 livres numériques lus par ce seul moyen. La plupart des plateformes de vente de livres numériques ont enregistré des hausses d'activité allant jusqu'à 200 %.

quelle politique votre ministère entend-il mener dans ce secteur d'activité d'importance pour notre pays, sur le plan tant culturel qu'économique ?

les contraintes et les obligations imposées par la crise sanitaire ont en effet favorisé une augmentation au moins temporaire des ventes et des prêts de livres numériques. Le développement du secteur du livre numérique est accompagné depuis plus d'une dizaine d'années par le ministère de la culture. Cela s'est manifesté notamment par l'adoption de la loi sur le prix unique du livre numérique en 2011, le soutien au développement du prêt numérique en bibliothèque ou encore le copilotage d'un plan stratégique pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles aux personnes en situation de handicap. En outre, le Centre national du livre (CNL) propose plusieurs dispositifs d'aide numérique, qui ont été refondus cette année. Trois aides sont dorénavant proposées afin d'accompagner la filière du livre dans le développement de services numériques structurants et interprofessionnels, de soutenir la publication et la diffusion de livres numériques, et de favoriser le développement du livre audio. L'imprimé demeure néanmoins le principal format du marché du livre, puisqu'il représente environ 95 % des ventes en volume. Les périodes de confinement liées à la crise sanitaire ont eu un impact sur les ventes, mais le soutien du Gouvernement a été important. Grâce à l'action du CNL et des directions régionales des affaires culturelles, le cas échéant en liaison avec les organismes de gestion collective et les collectivités territoriales, les différents maillons ont bénéficié d'aides variées. 677 auteurs ont reçu 2,26 millions d'euros d'aide d'un fonds d'urgence, et 440 aides ont été versées aux petites et moyennes maisons d'édition, pour plus de 4 millions d'euros. Les libraires ont en outre été soutenus à travers un fonds de compensation des pertes d'exploitation lors du premier confinement, pour plus de 15 millions d'euros. Le remboursement de leurs frais d'expédition pour leur permettre de poursuivre leur activité à distance lors du deuxième confinement a coûté plus de 3 millions d'euros.

À cela s'ajoutent les dispositifs transversaux que vous connaissez bien, et dont la chaîne du livre a pleinement bénéficié. Il faut conclure, madame la ministre. Combinée avec la fréquentation exceptionnelle des commerces de livres, l'action publique aura ainsi permis au secteur du livre de traverser avec le moins de dégâts possible la crise sanitaire.

à la hauteur de ces engagements que vous prenez pour défendre le livre. Puisse l'avenir vous donner raison

à la fois dans le Sahara algérien et en Polynésie française. En janvier dernier, vous preniez un décret créant une nouvelle agrafe « essais nucléaires », destinée à récompenser ces personnels par la médaille de la défense nationale. S'il s'agit d'une bonne nouvelle, c'est loin d'être suffisant, qu'il s'agisse des vétérans ou de leurs descendants. Les vétérans ne devraient-ils pas pouvoir bénéficier du statut d'ancien combattant ? N'ont-ils pas été exposés aux radiations nocives pour la santé en assurant l'indépendance stratégique de la France ? La demande qu'ils vous ont adressée à ce sujet, sauf erreur, n'a toujours pas obtenu de réponse. Ils sont nombreux à souffrir de lourdes séquelles dues à l'exposition aux rayonnements ionisants et à un environnement contaminé. Que leurs enfants et petits-enfants soient également touchés était également prévisible. Le lien entre l'exposition des vétérans et les conséquences néfastes sur leurs descendants a été démontré, et il est documenté depuis déjà un certain temps. Depuis Hiroshima et Nagasaki, on sait que l'irradiation des parents entraîne des conséquences irréversibles sur le génome : stérilité, malformations, cancers et autres pathologies apparaissent de génération en génération, ce qu'on observe également dans la lignée des vétérans des essais nucléaires français. Face à ce lourd tribut que payent les vétérans des essais nucléaires et leurs familles, le Gouvernement ne doit-il pas accorder aux descendants un suivi médical pris en charge par l'État ? N'y a-t-il pas là comme un devoir moral ? N'est-il pas de notre responsabilité d'assumer les conséquences des décisions prises dans le passé ? Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quand les demandes des vétérans

les vétérans des essais nucléaires par la médaille de la défense nationale. Cette distinction permet de récompenser les militaires d'active et de réserve, les anciens militaires ainsi que les civils qui justifient par tous moyens avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire. La mise en place de ce dispositif est très satisfaisante. Fin août, 1 145 médailles avec agrafe ont été décernées, et ce chiffre sera porté à 1 415 dans les prochaines semaines. L'État reconnaît ainsi ce qu'il doit à ces femmes et à ces hommes, qui se sont dévoués pour bâtir notre dissuasion nucléaire, pilier majeur de notre défense. En ce qui concerne le suivi sanitaire, je tiens d'abord à rappeler, en tant que médecin, toutes les précautions dont il faut s'entourer lorsqu'on aborde des données épidémiologiques.

médicale (Inserm) a rendu publique en 2021 l'expertise collective sur les effets sanitaires des essais nucléaires en Polynésie française. S'agissant des effets transgénérationnels ou héritables, cette expertise conclut que les études actuellement disponibles chez l'homme ne mettent pas en évidence d'effet décelable,

La commission internationale de protection radiologique a programmé une expertise sur les effets héritables des radiations, qui doit du comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants sont attendues pour 2028. Des experts de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribuent à ces travaux. Tout cela a été expliqué au cours des tables rondes que nous avons tenues les 1 et 2 juillet 2021, à la demande du Président de la République, avec nos amis polynésiens.

Merci, madame la ministre, pour votre réponse. J'attire toutefois votre attention sur la spécificité de ces essais nucléaires, qui devrait nous inviter à revoir la notion même d'ancien combattant,

les règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) entre communes demeurent toujours aussi injustes. Comme vous le savez, la part de la dotation forfaitaire par habitant varie du simple au double entre une commune rurale et une commune urbaine. Cette situation est totalement inacceptable et injustifiable. En effet, les études menées sur la réalité des charges supportées par les communes en fonction de leur taille montrent que la règle de calcul appliquée sous-estime les charges des communes de petite taille. Ce constat ancien a été confirmé par un rapport gouvernemental en 2020. Le Sénat a adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 un amendement qui réduisait cette inégalité. Malgré le caractère progressif et mesuré de cette proposition, la disposition a été supprimée à l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, ce dernier renvoyant à des réflexions complémentaires et ultérieures. Tout le monde s'accorde donc à dire qu'il faut revoir la règle, mais la situation demeure en l'état, comme en témoigne, malheureusement, le projet de loi de finances pour 2022, qui nous a été présenté la semaine dernière, puisque ce texte ne prévoit rien en la matière. Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, si, d'ici à l'adoption du projet de loi de finances pour 2022,

votre question porte sur un sujet auquel je sais le Sénat très attentif, celui des règles de répartition de la dotation forfaitaire entre communes. C'est une question sur laquelle circulent tout de même beaucoup d'interprétations erronées, et il faut redonner au sujet sa vraie portée, en rappelant que ce coefficient sert uniquement à traduire dans l'attribution des aides de l'État le fait que les communes, en règle générale, supportent d'autant plus de charges qu'elles comptent d'habitants.

ont reçu 166 euros de dotation par habitant, contre 160 euros pour les communes rurales. En effet, au-delà de la dotation forfaitaire, dans le calcul de laquelle joue le coefficient logarithmique, les communes rurales reçoivent aussi d'autres aides. Je pense en particulier à la dotation de solidarité rurale, dont le montant s'élève à 1,8 milliard d'euros. Cette année encore, le Gouvernement propose d'augmenter cette dotation de 95 millions d'euros dans le projet de loi de finances, ce qui portera à 455 millions d'euros sa progression depuis le début du quinquennat. Je pense aussi à la qui s'élèvera toujours à 1,46 milliard d'euros en 2022, ce qui fait 5,2 milliards d'euros sur ce quinquennat contre 3,5 milliards d'euros sous le précédent. En ce qui concerne les évolutions que vous appelez de vos voeux,

villes moyennes, petites villes ou grands centres urbains -, car le Gouvernement ne souhaite pas réformer la DGF contre la volonté des élus et sans esprit de consensus. Le président du comité des finances locales a d'ores et déjà indiqué que les travaux du groupe, qui se poursuivent depuis deux ans, se prolongeront en 2022. Je crois qu'il faut saisir cette opportunité pour en débattre sereinement et surtout de façon coordonnée,

Madame la ministre, je suis assez étonné par votre réponse. Vous commencez par expliquer que, finalement, tout cela est très justifié, ce qui est tout de même assez surprenant, parce que, jusqu'alors, on avait plutôt entendu les membres des gouvernements précédents reconnaître qu'il y avait un vrai problème et qu'il fallait se pencher dessus. Là, vous nous dites finalement de circuler, qu'il n'y a rien à voir, et qu'il n'est pas gênant que la dotation forfaitaire varie du simple au double en fonction de la taille de la commune. C'est une nouveauté, j'en prends acte, le Sénat en prend acte et je suis certain que les maires ruraux apprécieront et qu'ils en prendront acte également. Dans le même temps, vous nous dites tout de même qu'on va continuer à réfléchir, jusqu'en 2022 ... C'est ce qu'on nous dit chaque année. Pour être très direct avec vous, donne, une fois de plus, le sentiment d'être menés en bateau, ce qui est extrêmement désagréable pour les nombreux élus concernés. Le Sénat, une fois de plus, évoquera ce sujet lors de la discussion du prochain projet de loi de finances en espérant- on peut toujours espérer -être enfin entendus par le Gouvernement !

Ces prestations sont soumises à conditions de ressources. L'indemnité de fonction de l'élu entre en compte dans le calcul de ses ressources et peut être cumulée avec ces prestations, dans la limite du dernier salaire annuel moyen perçu avant leur attribution. En l'état actuel des choses, il n'y a pas formellement d'interdiction de cumuler une pension d'invalidité et une indemnité de fonction, mais il y a un plafonnement du cumul des ressources susceptibles d'être procurées par l'addition de l'une Il existe même, implicitement mais clairement, une autorisation de cumul lors des six premiers mois de la reprise d'une activité- du mandat, en l'occurrence -, puisque ce n'est éventuellement qu'à l'expiration de ces deux trimestres que la pension sera suspendue ou supprimée. supprimée. Franchement, cela crée une inégalité de fait entre élus et n'incite pas les personnes en situation d'invalidité ou du handicap à s'engager dans la vie politique. En pratique, l'addition des deux ressources conduit souvent l'élu local à dépasser le plafond ou à devoir faire un choix.

Je vous remercie excède le salaire antérieur à l'attribution de la pension d'invalidité, tout revenu gagné au-delà de ce seuil se traduit par une réduction à due concurrence du montant de la pension d'invalidité. Mais cette règle ne concerne pas seulement les élus. Elle s'applique également pour tous les revenus d'activité. Je pense qu'elle soulève une difficulté beaucoup plus large. Alors que près de 31 % des bénéficiaires d'une pension d'invalidité travaillent, l'application de ces règles de cumul constitue une forte désincitation

C'est pourquoi nous avons annoncé un assouplissement des règles de calcul entre pensions d'invalidité et revenus d'activité dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Cette réforme prévoit un cumul intégral des revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le revenu disponible de l'assuré redevienne similaire à celui qu'il avait avant son passage en invalidité, de la même façon qu'aujourd'hui. Mais, au-delà de ce seuil, la pension d'invalidité ne sera réduite que de la moitié des gains constatés, ce qui supprimera l'effet couperet actuel. Cette réforme s'appliquera également dans les mêmes conditions aux indemnités perçues par les élus locaux. Elle facilitera le maintien dans l'emploi de ses assurés, mais aussi l'exercice d'un mandat électoral en maintenant un gain financier pour tout revenu supplémentaire. Elle doit être mise en oeuvre par un texte réglementaire en cours de finalisation et interviendra au printemps 2022. Je crois, madame la sénatrice, qu'une telle réforme répondra aux difficultés que vous avez soulignées tout en garantissant une équité de traitement entre les différents types de revenus perçus par les pensionnés d'invalidité.

n'est pas un salaire ! Je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence entre des personnes à la retraite, des personnes au chômage ou des personnes en activité, qui peuvent percevoir l'intégralité de leurs indemnités,

et de la relance. Monsieur le secrétaire d'État, depuis le début de l'année, les acteurs français de la filière bois sont confrontés à d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières. Plusieurs essences destinées à la construction et à des usages nobles sont concernées par ce phénomène, comme le chêne, le hêtre, les résineux ou le douglas du Morvan. Ces difficultés s'expliquent par les exportations massives de grumes vers l'Asie. Les expéditions de bois brut issu de forêts françaises se font plus particulièrement vers l'économie chinoise, qui connaît une forte reprise depuis plusieurs mois. Ces bois bruts expédiés par containers font défaut aux scieries françaises. Ainsi, 90 % des scieries de chênes n'ont plus assez de bois pour assurer leurs besoins de l'année. Dans ce contexte, des constructeurs de maisons en ossature bois situés dans le Morvan sont confrontés à un doublement des prix de la matière première ou ne trouvent carrément plus de bois pour poursuivre leur activité. Ce phénomène s'étend également au volume de résineux avec des acheteurs étrangers qui perturbent leurs achats. Cette situation difficile s'est accélérée et amplifiée avec la décision de la Russie de bloquer ses exportations de grumes et de sciage auprès de son client principal, l'Asie. Dans ce contexte, l'industrie française du sciage et de la deuxième transformation se trouve en grand danger, avec le ralentissement, voire l'arrêt de ses activités. C'est d'autant plus regrettable que la reprise économique est bien présente. À cela s'ajoute le gâchis écologique que constituent les exportations de grumes depuis les forêts françaises vers l'Asie. Ces expéditions ont pour conséquence d'annuler le bénéfice de la captation du carbone par le bois. Monsieur le secrétaire d'État, comme vous le savez, la filière du bois occupe une place particulièrement importante dans l'économie de nos régions, en particulier dans le Morvan.

Ces dynamiques ne sont pas sans risques pour la filière : elles peuvent entraîner des hausses de coût, des augmentations de délais, voire des pénuries en bois brut. La capacité de nos industries à être présentes sur le marché du bois de construction en plein essor est d'ailleurs une question de souveraineté. Pour résorber ces tensions d'approvisionnement, le Gouvernement a saisi la Commission européenne en lui demandant de prendre des mesures de sauvegarde au titre de la compétence commerciale et d'éviter ainsi l'emploi sous-optimal des ressources forestières européennes. Le Premier ministre a aussi demandé à l'Office national des forêts de développer au maximum les contrats d'approvisionnement avec les scieries françaises, pour éviter que la production de bois des forêts domaniales ne soit vendue aux enchères, s'exposant ainsi à l'action de traders qui exportent souvent hors d'Europe. Dans le cadre du plan France Relance, le Gouvernement va également redéployer 100 millions d'euros supplémentaires pour abonder les différents dispositifs de soutien à la filière forêt et bois. Ils s'ajoutent donc aux 200 millions d'euros déjà consacrés à la relance de la filière : 150 millions d'euros pour le renouvellement forestier en amont- cela correspond au reboisement de 45 000 hectares, soit environ 50 millions d'arbres -et 50 millions d'euros pour la modernisation des industries de transformation du bois en aval. Enfin, pour assurer l'avenir à long terme de cette filière d'importance nationale et si particulière pour notre société, le Premier ministre a demandé aux ministres Julien Denormandie, Agnès Pannier-Runacher et Bérangère Abba d'organiser à l'automne des assises de la forêt et du bois. Elles doivent être un espace de dialogue, décliné dans les territoires, en cohésion avec les acteurs amont et aval, mais aussi les experts et les associations, pour nourrir la vision la plus large possible de la forêt française et de la filière bois de demain. Elles permettront de partager les enjeux du patrimoine forestier que nous avons en commun, pour que nous puissions collectivement faire prospérer cette richesse. La parole

Cette cession consiste à créer une nouvelle entité, dont l'autonomie est prévue en 2022, rassemblant des activités commerciales et de développement de principes actifs pharmaceutiques de Sanofi, et six de ses sites de production en Europe. D'après les représentants du personnel, cette cession illustre la stratégie de « vente à la découpe » de Sanofi, le démantèlement futur du groupe et un recul fort de son empreinte industrielle en France. L'avenir des deux sites français- le deuxième étant situé à Elbeuf, en Seine-Maritime -dans ce nouvel ensemble inquiète les employés, qui souhaitent préserver l'outil de production et les emplois. En effet, l'état de vétusté des équipements des sites français, qui pénalise la performance de manière systémique, tout comme l'augmentation continue des coûts de revient industriels, nécessite des investissements lourds. Malgré l'annonce rassurante d'EuroAPI début septembre de la construction d'un bâtiment pour la production d'hormones, moyennant un investissement de 50 millions d'euros, quelques inquiétudes persistent. L'enjeu est majeur pour ce secteur rural du Puy-de-Dôme : le site Sanofi de Vertolaye compte 630 salariés en CDI et 100 à 150 contrats temporaires. On arrive à environ 1 000 emplois avec les différents partenaires. Outre l'enjeu d'aménagement du territoire, il s'agit d'un sujet d'intérêt général sur la capacité de l'industrie pharmaceutique française à produire des médicaments pour la santé de nos concitoyens et à éviter de nouvelles ruptures de médicaments essentiels, voire vitaux. La crise sanitaire que nous traversons toujours nous a douloureusement rappelé le constat de perte d'autonomie de la France dans la production industrielle et ses conséquences néfastes. Le Président de la République a annoncé en juin 7 milliards d'euros de crédits pour l'innovation en santé, 1 milliard d'euros étant déjà programmés pour le secteur du médicament dans le budget 2022. Ce sont des investissements massifs, qui doivent se concrétiser par un soutien et un renforcement des entreprises déjà présentes sur nos territoires. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous rassurer sur l'avenir d'EuroAPI en France et la pérennité de l'industrie pharmaceutique sur le site de Vertolaye ? La parole

vous l'avez dit, la crise sanitaire a montré que nous devons plus que jamais avoir des industriels de la santé forts, résilients et capables de faire face à la concurrence mondiale, qui est toujours plus forte. Le 24 février 2020, Sanofi a annoncé la cession d'une partie de ses activités de chimie pharmaceutique en Europe, visant six sites industriels européens, dont deux sites français : Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Vertolaye. La société issue de cette opération, EuroAPI, a pour objectif de devenir le leader européen de la production de principes actifs, au deuxième rang mondial, derrière le suisse Lonza. Cette entreprise possédera des atouts, en particulier un large portefeuille de produits, des normes de qualité élevées, des prix compétitifs sur le marché des produits à forte valeur ajoutée, des capacités industrielles et technologies de pointe dans toute l'Europe, et un réseau commercial présent dans plus de 80 pays. Sur les modalités de création d'EuroAPI, le Gouvernement a demandé à Sanofi plusieurs garanties auxquelles s'est engagée l'entreprise : l'empreinte industrielle et les emplois de Sanofi sur le territoire français seront garantis, avec 1 500 emplois sur les 3 200 salariés de la nouvelle entité qui seront en France EuroAPI aura son siège social en France, à Paris ; et Sanofi restera un actionnaire de référence, avec 30 % du capital. Le site de Vertolaye, dans le Puy-de-Dôme, et ses près de 800 collaborateurs apporteront à EuroAPI toutes leurs capacités dans la fabrication de principes actifs. notamment reconnu en Europe pour son expertise en procédés chimiques complexes et sa production d'anti-inflammatoires. Fin août, la direction d'EuroAPI a annoncé la construction d'un nouveau bâtiment « Hormones » sur le site de Vertolaye à l'horizon 2023. Ce projet a pour objectif d'assurer la continuité de l'expertise et du savoir-faire de Vertolaye sur la fabrication de produits hautement actifs. Un investissement de l'ordre de 40 à 60 millions d'euros permettra la construction de ce nouveau bâtiment, à la pointe des outils disponibles à l'heure actuelle. Un plan d'investissement de 190 millions d'euros a été annoncé par ailleurs sur le site de Vertolaye à l'horizon 2025. Dans le cadre du dialogue social interne, des réunions avec les représentants du personnel ont été organisées pour accompagner la mise en place de ce projet et expliquer l'opportunité qu'il représente dans un contexte post-covid. Le Gouvernement demeure très attentif aux choix et à la stratégie industrielle de Sanofi. Les investissements étrangers dans EuroAPI devront à ce titre être soumis à la procédure des « investissements étrangers en France », car les activités d'EuroAPI relèvent de secteurs stratégiques. J'ajoute que, dans le cadre du futur plan d'investissement qui doit être présenté dans les jours à venir par le Président de la République,

secrétaire d'État, permettez-moi d'insister de nouveau sur la nécessité de préserver les emplois, donc sur Vertolaye, mais aussi sur l'importance de ce site pour le département du Puy-de-Dôme et pour l'industrie pharmaceutique française et son autonomie

il y a un an, dans le cadre des accords du Ségur de la santé, beaucoup déploraient l'absence du secteur de l'aide à domicile des mesures de revalorisation salariale des métiers difficiles. Cet oubli avait été ressenti de façon très injuste, d'abord par les acteurs eux-mêmes, dévoués et aux prises avec de véritables difficultés, mais aussi par tous ceux qui ont pris les devants, comme les conseils départementaux, qui avaient institué des primes. Dans cette crise, de nombreuses initiatives ont été prises sur le terrain. Les critiques ont porté, et j'en suis heureuse. On a ainsi annoncé la refonte de l'avenant 43, avec une refonte complète de la grille conventionnelle destinée à augmenter le salaire des personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ainsi que ceux des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad). Cette augmentation doit entrer en vigueur au 1 octobre 2021. On annonce également que l'État contribuera à hauteur de 200 millions d'euros annuels au financement des conseils départementaux. Ces décisions sont certes heureuses, mais elles auront un impact majeur sur les conseils départementaux. Et il ne suffit pas de réagir sur le coup, car il y a un trou dans les mesures de revalorisation. Il faut aussi réfléchir à long terme et voir plus en amont les problèmes de recrutement qui se poseront. Peut-on réagir par du simple saupoudrage ?

Révélé par la crise, l'engagement de ces professionnels les honore. C'est un métier noble, souvent exercé par des femmes à temps partiel, qui mériterait davantage de reconnaissance, à l'exemple de la prime covid, dont j'ai obtenu le financement dès mon arrivée à l'été 2020. Seuls

pour accompagner le souhait massif de nos concitoyens de vivre à domicile le plus longtemps possible, même lorsqu'une perte d'autonomie les atteint. Il fallait donc apporter une première réponse aux salariés de la branche de l'aide à domicile. Ils l'attendaient. Ils ont ouvert des négociations conventionnelles, et j'ai agréé leurs accords l'été dernier. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a permis de faire en sorte que l'État accompagne le financement de cette revalorisation, qui entrera en vigueur dans trois jours. Le coût de cette revalorisation pour les départements, qui en assument la compétence, sera allégé de moitié, et même de 70 % en 2021. C'est historique, tant par les montants mobilisés que par la démarche partenariale. Mais vous avez raison, cela ne concerne que les aides à domicile exerçant dans un réseau associatif. Nous avons besoin d'accompagner toutes les

C'est pourquoi, comme le Premier ministre l'a annoncé jeudi dernier, il sera proposé au législateur de créer un tarif plancher national applicable par tous les départements pour revaloriser du handicap). Cette disposition sera portée dans le cadre du prochain PLFSS, avec un montant pour ce tarif socle de 22 euros par heure applicable à partir du 1 janvier 2022, garanti par un financement d'État pérenne.

qui exercent dans nos stations de sports d'hiver françaises et répondent aux besoins de soins des populations, s'agissant notamment de la traumatologie liée à la pratique des sports d'hiver, au premier rang desquels figure Cette spécificité nécessite un plateau technique adapté en radiologie, échographie, médecine d'urgence et petite chirurgie, faisant ainsi de ces cabinets médicaux de véritables petites cliniques de proximité, qui évite de nombreux transports et passages dans les services d'urgence des hôpitaux en vallée, souvent situés à une heure de route. La spécificité de ces cabinets médicaux réside à la fois dans les frais fixes particulièrement élevés liés à ces équipements de pointe et à la grande saisonnalité de leur activité. Or, depuis le début de la crise sanitaire et la non-ouverture des domaines skiables durant l'hiver 2020-2021, les cabinets médicaux de montagne ont accusé une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 58 %. Sous la pression des élus de la montagne, le Gouvernement a corrigé le dispositif d'indemnisation des médecins « DIPA 3 », qui se réfère aux revenus mensuels, en lieu et place de la moyenne annuelle des revenus, afin de prendre en compte cette saisonnalité. Or il s'avère qu'au niveau local les CPAM n'auraient à ce jour pas eu connaissance de ce changement de méthode de calcul, privant ainsi les médecins de montagne des compensations promises et fragilisant un peu plus leur situation.

Ce dispositif a pour objectif d'aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans le contexte que vous présentez. Le Gouvernement a souhaité réactiver ce DIPA à plusieurs reprises pour tenir compte, chaque fois que cela était nécessaire, des pertes d'activité subies par certains professionnels se trouvant dans des situations particulières. Il a en particulier été réactivé pour les professionnels de santé installés dans les zones de montagne pour la période du 1 décembre 2020 au 30 avril 2021, en raison de l'impact sur leur activité de la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski. Vous l'avez rappelé, les professionnels qui y exercent ont une fluctuation assez forte de leurs revenus, compte tenu de la saisonnalité C'est pourquoi il a été prévu que l'aide accordée aux professionnels qui exercent en montagne, dans des territoires concernés par cette spécificité, prenne en compte, à la différence des autres DIPA, la saisonnalité de leurs revenus. Le dispositif est conçu en deux temps. professionnels ont pu, dès son instauration, solliciter une avance sur la base d'un calcul prévisionnel de l'aide. Néanmoins, cette aide prévisionnelle est simulée sur le téléservice sur le téléservice général, sans prendre en compte la saisonnalité propre au dispositif Montagne. Il était nécessaire de s'appuyer sur le dispositif existant afin de s'assurer d'un versement rapide des avances. La saisonnalité sera bien prise en compte par le versement d'une régularisation dès que sera calculé, pour dès que sera calculé, pour chaque professionnel, le montant définitif de son aide. Elle sera ainsi indexée aux revenus des mois équivalents des années précédentes. Les paramètres précis de cette saisonnalité seront communiqués en amont, tant aux professionnels qu'à leurs caisses primaires d'assurance maladie. l'État tiendra son engagement d'un accompagnement spécifique des professionnels de santé exerçant en montagne. madame la ministre. J'espère vraiment que tout cela se traduira concrètement sur le terrain, car les professionnels de santé sont actuellement assez inquiets. est vraiment nécessaire de les sauvegarder, car ils jouent un rôle très important dans nos territoires. En haute saison touristique, il n'est pas rare que la population y soit multipliée par dix.

de la santé. Madame la ministre, la crise sanitaire a eu un impact terrible sur la santé psychologique de tous nos compatriotes. Le Président de la République l'a lui-même reconnu. Il a annoncé la mise en place de dix consultations gratuites chez un psychologue pour les mineurs âgés de 3 à 17 ans qui le souhaitent. Cette mesure est utile pour lutter contre les effets dévastateurs de la crise sanitaire sur la santé physique et mentale de nos concitoyens. Les adultes aussi sont touchés par ce fléau. Certains pays voisins ont mis en place des solutions efficaces. En Suisse, des infirmières psychiatriques libérales sont envoyées au domicile des personnes vulnérables par des psychiatres pour évaluer la santé mentale de leurs patients et les accompagner. La France devrait à mon sens suivre cet exemple et comptabiliser ces suivis à domicile comme des soins pour que les infirmières libérales soient rémunérées à leur juste valeur. Madame la ministre, le Gouvernement entend-il expérimenter de telles mesures ?

constante du Gouvernement, et j'en veux pour preuve les assises nationales de la santé mentale, qui se tiennent depuis hier, et qui seront conclues par le Président de la République. Classés au premier rang des maladies en termes de dépenses de soins, avant même les cancers et les maladies cardiovasculaires, les troubles psychiques et leur prise en charge représentent un enjeu majeur, d'autant qu'ils affectent près d'un quart des Français. Le besoin est de surcroît précoce, puisque 15 % des 15-20 ans auraient besoin d'un suivi ou de soins. C'est indéniable, la dégradation de la santé mentale des Français a constitué un lourd tribut payé pour nous permettre de surmonter la pandémie de covid-19. Le suivi renforcé de la santé mentale des Français, organisé par Santé publique France, illustre que les états anxieux ou dépressifs, les problèmes de sommeil se sont accrus pendant la crise, avec une augmentation des passages aux urgences et hospitalisations pour les plus jeunes. Pour y répondre, le Gouvernement s'est engagé fermement. D'abord, en rappelant toujours qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Dès le mois d'avril 2021, une campagne grand public a été lancée : « En parler, c'est déjà se soigner. » Elle a permis de diminuer la stigmatisation des personnes souffrant de troubles et faciliter le recours aux soins et à la prévention. Ensuite, les expérimentations lancées dans le cadre de la feuille de route Santé mentale et psychiatrie et les dispositifs d'urgence existants mis en place pendant la crise ont, à l'épreuve de cette crise, montré l'intérêt d'un repérage et d'une prise en charge précoces des troubles psychiques légers à modérés. La CNAM expérimente la prise en charge par des thérapies non médicamenteuses pour les adultes. Nous poursuivons l'expérimentation Écout'Émoi, destinée aux jeunes en détresse psychologique, et nous maintenons les dispositifs d'urgence PsyEnfantAdo et SantéPsyEtudiant, mis en place en période de crise sanitaire. Enfin, vous savez que nous avons renforcé les centres de santé et maisons de santé en psychologues, le Ségur de la santé, permettant ainsi une proximité accrue, sur le modèle que vous semblez proposer. Les assises de Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie sont au coeur de ce constat. Elles ont vocation à aller plus loin, pour en finir avec le tabou sur la santé mentale. Des annonces devraient être faites en ce sens dans la journée. La parole

de la santé. Madame la ministre, je voudrais attirer votre attention sur la situation des malades atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot. Cette maladie, décrite il y a plus de 150 ans, touche des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Environ 2 000 personnes sont diagnostiquées atteintes de SLA en France chaque année. Il n'y a malheureusement aucun traitement, et la maladie reste toujours mortelle, avec un délai moyen de survie de trois Beaucoup de recherches ont lieu partout pour comprendre la pathogenèse de cette maladie de Charcot, sans que l'on ait aujourd'hui de cause précise, tout au plus un ensemble de facteurs, y compris une sensibilité génétique, qui concourent à l'apparition des symptômes. Un certain nombre d'études portent sur le rôle du microbiote intestinal, qui serait perturbé dans bon nombre de cas, d'où l'idée d'un transfert d'un microbiote sain à ces patients. Une association, Tous en selles contre la SLA, étudie le lien entre un axe cerveau-intestin et cette pathologie neurodégénérative. Elle propose une transplantation de matières fécales, aussi appelée greffe fécale, de selles humaines d'un sujet sain à un patient touché par une altération du microbiote comme dans la SLA. Les patients pourraient voir leurs symptômes atténués et continuer à vivre dans de meilleures conditions de confort. (ANSM) précise qu'en l'absence d'un rapport bénéfice-risque clairement établi cette thérapie doit être réservée aux situations graves ou rares, en échec de traitement conventionnel et en l'absence d'alternative thérapeutique disponible et appropriée. C'est le cas de la SLA, pour laquelle aujourd'hui aucun traitement n'apporte de modifications de l'évolution de la pathologie ni de confort au patient. Pour le comité scientifique FilSLAN, mettre à disposition la thérapie sous forme de délivrance à titre compassionnel serait possible sous réserve de l'accord de l'ANSM.

thérapeutiques et entend le rester, en accompagnant au mieux le développement de cette thérapie. La transplantation de ce microbiote a donné de premiers bons résultats comme traitement du Clostridium difficile et suscite de nombreux espoirs pour traiter d'autres pathologies comme la dysbiose intestinale. Après vérification auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), plusieurs essais cliniques ont été autorisés en France pour des indications en lien avec la maladie de Crohn. La maladie de Charcot ne figure en revanche pas parmi les indications validées ou en cours de validation dans notre pays, à ce stade. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt « Nouvelles biothérapies et outils de production », lancé début 2021 par Bpifrance, plusieurs projets impliquant l'utilisation de microbiote fécal ont été reçus et sont en cours d'instruction. Leurs applications thérapeutiques sont l'oncologie, la maladie de Crohn, le diabète et l'obésité liés à la stéatose hépatique. Les services du ministère de la santé n'ont cependant pas connaissance de projets dont l'application thérapeutique serait la maladie de Charcot. La réforme de l'accès précoce

dans une indication thérapeutique donnée, au titre de l'accès compassionnel. Cette autorisation ne pourra être octroyée que si le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans l'indication considérée, s'il n'existe pas de traitement approprié et si l'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles. La demande d'autorisation est sollicitée par le prescripteur pour un patient nommément désigné. Par ailleurs, certaines pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé peuvent, dans certaines conditions, réaliser des préparations en vue de la transplantation de microbiote fécal

Ainsi, les professionnels des établissements publics autonomes d'Eure-et-Loir ne sont pas concernés par la mise en oeuvre du complément de traitement indiciaire (CTI). Or, tout comme leurs collègues des hôpitaux ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ils relèvent de la fonction publique hospitalière et sont soumis aux mêmes obligations de service. Ils sont restés pleinement mobilisés pendant la pandémie. L'équité de traitement entre les agents concernés semble rompue sans que cela soit justifié. De surcroît, cette différence de traitement entraînera de nouvelles difficultés les établissements non concernés par le CTI subiront la concurrence des établissements qui le proposent lorsqu'ils recruteront à des fonctions similaires. La qualité des accompagnements pâtira de cette concurrence entre établissements. L'attribution du CTI doit impérativement concerner l'ensemble des professionnels, chacun oeuvrant, par son métier, à l'accompagnement des jeunes et des adultes en situation de handicap. Au regard de l'unité du statut de la fonction publique hospitalière, il conviendrait d'étendre l'éligibilité au CTI à toutes les catégories de personnels du social et du médico-social.

le 1 juin 2021 d'une augmentation salariale. Ces discussions se sont poursuivies avec les organisations syndicales au sujet des professionnels des établissements médico-sociaux publics autonomes. Ces travaux ont abouti à un nouveau protocole, signé le 28 mai dernier, qui étend le bénéfice du CTI à l'ensemble des personnels soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, titulaires et contractuels de ces structures financées pour tout ou partie par l'assurance maladie, à compter du 1 octobre 2021.

Certains établissements ont fait l'objet de négociations compte tenu de leur proximité avec le parcours de soins à l'hôpital ou en Ehpad. Dans d'autres secteurs, toute revalorisation ne peut se faire que dans le cadre d'une discussion approfondie avec les collectivités dont dépendent ces politiques. Le Gouvernement fait preuve de volontarisme pour apporter une réponse pérenne et surtout équitable à ces professionnels, dans le respect des compétences dévolues à toutes les parties.

En 2019, la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, chargée d'évaluer l'intérêt thérapeutique de ces produits dans le panier de soins remboursables, soulignait l'existence de différents traitements actuellement pris en charge dans le traitement de fond de la migraine, pouvant être considérés comme des comparateurs cliniquement pertinents de ces nouvelles spécialités. Ces comparateurs permettent une prise en charge de l'ensemble des stades de la pathologie avec des traitements de première et seconde intention - comme le Lopressor ou le Seloken mais également des traitements de recours - comme le Nocertone ou le Sibelium -, ainsi que des alternatives non médicamenteuses. C'est pourquoi la Haute Autorité de santé recommande la prise en charge de ces traitements par la solidarité nationale pour les seuls patients

Comme vous le savez, la loi prévoit que la fixation du prix d'un médicament tient compte de l'amélioration du service médical rendu par le médicament. Les discussions tarifaires entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les laboratoires exploitant ces spécialités se sont ainsi fondées sur les critères légaux, réglementaires conventionnels en vigueur. Une spécialité d'ASMR 5 ne peut être inscrite au remboursement que dans le cas où elle permet de diminuer les coûts des traitements fait plusieurs propositions aux laboratoires, ces discussions n'ont pu aboutir du fait des prétentions tarifaires extrêmement élevées des industriels concernés au regard des dépenses actuellement engagées pour le traitement médicamenteux de la migraine. L'échec des négociations tarifaires n'a pas permis d'inscrire cet antimigraineux sur les listes des médicaments remboursables. Pour autant, le ministère, sous l'impulsion d'Olivier Véran, continue d'engager des travaux pour renforcer l'expertise scientifique sur ce sujet. De nouvelles négociations pourraient avoir lieu si le laboratoire se montre ouvert à la discussion ou présente des éléments tangibles à la commission de la transparence.

la protection sociale de l'ensemble des Français, supporte pour les tests antigéniques, ainsi que pour les vaccins. Comment tout cela est-il financé ?

Canévet, votre question est claire, elle porte non pas sur l'opportunité médicale de l'action que nous avons menée, mais sur le coût des tests et des vaccins, ainsi que sur l'accompagnement des collectivités. Monsieur le sénateur, je pense qu'il manque toujours à ces données, lorsqu'on les évoque, le coût de l'absence de soins, le coût social, sanitaire et économique d'un non-choix.

Ces derniers ont un coût unitaire de 43,89 euros, auquel peut s'ajouter un bonus si le résultat est rendu en moins de douze heures. Ces informations sont régulièrement communiquées par le Gouvernement ; vous vous êtes d'ailleurs appuyé sur elles pour formuler votre question. Sur les 14,8 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles engagées par l'assurance maladie en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire, 6,2 milliards sont dédiés au financement des tests de dépistage, qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Compte tenu de l'évolution de la crise et de l'avancée de la campagne de vaccination, les tests cesseront d'être pris en charge intégralement par l'assurance maladie au 15 octobre 2021. Ils resteront remboursés pour raison médicale, sans prescription pour les personnes déjà vaccinées, sur prescription pour les autres.

À cela s'ajoutent les achats de vaccins eux-mêmes, réalisés par Santé publique France, et qui font l'objet de contractualisations fortes, nécessaires pour faire face aux retards que nous avons connus. Je ne dispose donc pas à ce jour du montant consolidé de ces achats. Enfin, vous avez raison de souligner l'importance du rôle joué par les collectivités

La carte de la vaccination est aussi celle de la précarité sociale. Pour tenter de résoudre ce problème du moindre recours à la vaccination, des villes ont mobilisé des moyens très importants. Je pense à la ville de Bagneux, dont je suis l'élu, qui a consacré près de 400 000 euros à son centre de vaccination. Le Gouvernement ne lui a apporté qu'une aide symbolique de 76 000 euros Malgré ces efforts importants, de nombreuses populations demeurent rétives à la vaccination. Ce ne sont pas les mesures coercitives, comme le passe sanitaire, qui les inciteront à se faire vacciner, car ces personnes n'ont souvent qu'une vie sociale réduite, simplement destinée Depuis trois mois, la Croix-Rouge de Bagneux, avec l'aide de la ville, a mis en oeuvre des centres de vaccination ambulatoires au plus près des populations. J'ai visité samedi 11 septembre celui qui est installé place Dampierre. Ouvert de huit heures à dix-huit heures, il a permis de vacciner 111 personnes, dont 39 ont reçu une première dose.

Il est toujours plus facile d'accepter la vaccination quand c'est votre voisin qui vous la propose. Ce centre va s'installer dans d'autres quartiers de Bagneux.

Monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias, j'ai moi-même aussi sillonné tous les centres de vaccination à travers la France, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. J'ai vu toutes les initiatives intéressantes prises partout sur le territoire français. Les collectivités territoriales ont été au rendez-vous.

Votre question est posée dans un contexte d'évolution de cette campagne vaccinale puisque nous devons, d'une part, assurer les rappels pour les personnes éligibles et, d'autre part, accroître davantage le taux de primo-vaccination. parvenir, nous devons atteindre des publics assez hétérogènes, vous en conviendrez. Il s'agit souvent de jeunes résidant en périphérie de grandes métropoles, de personnes âgées isolées, ou encore de personnes en situation de grande précarité financière.

Nous avons ouvert des créneaux de vaccination sans rendez-vous, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Nous nous sommes assurés que tous les centres d'hébergement d'urgence avaient reçu la visite d'au moins une équipe pour proposer la vaccination à leurs résidents. Des navettes ont été mises en place pour conduire les personnes dans les centres de vaccination, des « vaccibus » et « vaccicars » ont été déployés pour informer la population

de la santé. Madame la ministre, la crise sanitaire de la covid-19 a affecté tous les secteurs de la santé, plus particulièrement celui de la psychiatrie. L'enjeu est majeur, puisque l'on estime qu'une personne sur cinq sera potentiellement atteinte d'une maladie psychiatrique. Les confinements successifs, conjugués aux difficultés économiques et sociales, ont eu pour effet d'augmenter les syndromes dépressifs, anxieux et les addictions. Cette situation a engendré de nouveaux besoins en matière de santé mentale. Avant même le début de la crise sanitaire, le contrôleur général des lieux de privation de liberté se faisait l'écho des nombreuses difficultés des établissements de santé mentale, au premier rang desquelles figurait la suroccupation constante, la pénurie de personnel soignant compétent ne permettant pas aux établissements d'offrir une même qualité de prise en charge. cas, la prise en charge reste insuffisante. En dépit du professionnalisme et de la remarquable adaptabilité dont fait preuve le personnel soignant, les confinements successifs ont évidemment la situation. Durant cette même période, nombre de structures extrahospitalières, notamment les hôpitaux de jour, ont dû fermer. Dans son dernier rapport d'activité publié au mois de juillet 2021, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé que, durant cette période, à défaut de directives de portée nationale, la situation a été gérée sur le fondement de décisions locales, avant qu'une concertation ne se mette en place autour des structures qui pilotent la psychiatrie au quotidien. Cela n'a pas été sans conséquence pour les patients qui, dans ce contexte, ont subi des restrictions excessives de leurs droits. Ainsi, il n'est pas surprenant de constater que, après le confinement, les services de santé mentale aient vu affluer des patients ayant renoncé à leurs soins pendant cette période, leur pathologie s'étant parfois aggravée. Face à une crise inédite, à laquelle s'ajoute la mutation de la patientèle et de la demande collective, tout concourt au découragement et à l'épuisement des professionnels de la filière psychiatrique et à une baisse de la qualité et de l'efficacité des soins.

vous l'avez rappelé, en ce moment même se déroule la deuxième journée des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. S'il était besoin de démontrer l'intérêt que nous portons à cette question, ces Assises parlent

ces Assises vont permettre aux professionnels, aux patients, à leurs familles, ainsi qu'à tous les citoyens de s'informer et de débattre des sujets de santé mentale et de psychiatrie dans leurs grandes orientations. J'ai eu l'honneur de conclure hier la première journée de ces Assises. J'ai été particulièrement impressionnée par la qualité des intervenants et des interventions, ainsi que par la pluralité des thématiques abordées. Je suis convaincue que ces Assises marqueront une étape clef et permettront d'avancer vers une meilleure prise en charge de la santé mentale des Français.

Nous avons soutenu financièrement les établissements de psychiatrie : 110 millions d'euros de crédits pérennes supplémentaires ont été octroyés aux établissements de psychiatrie publique par une dotation annuelle de financement en 2020 et en 2021. C'était l'une des priorités fixées dans la feuille de route de la psychiatrie et de la santé mentale. Les appels à projets nationaux mis en place depuis 2019 concernant le fonds d'innovation en psychiatrie et en pédopsychiatrie ont été reconduits en 2020 et en 2021 afin de renforcer l'offre de psychiatrie et la qualité des soins aux patients. Ils ont permis, notamment, la création de lits dans les territoires les plus dépourvus, en particulier pour proposer des conditions adaptées à l'hospitalisation des mineurs. Le Ségur de la santé renforce les centres médico-psychologiques (CMP) et les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) en psychologues. La revalorisation salariale et l'exercice mixte en ville et à l'hôpital contribueront à l'attractivité de cet exercice pour les psychiatres.

concret : la compensation par l'État des surcoûts liés à la vaccination. En effet, madame la ministre, les élus locaux dans les Alpes-Maritimes, comme sur l'ensemble du territoire, ont été de nouveau au rendez-vous, en augmentant la capacité des centres de vaccination au gré des annonces gouvernementales. L'État s'était engagé à compenser les dépenses associées. Aujourd'hui, la compensation promise, quand elle existe, est loin de couvrir les coûts réels. Elle correspond à peine à un pourboire. est la réalité de nos territoires : des collectivités que nous envoyons au front avec leurs propres moyens, un président plus prompt, en cette période, à ouvrir le carnet de chèques qu'à honorer cette dette,

en mettant à disposition de la campagne vaccinale, pour leurs administrés, des membres de leur personnel et des locaux. Aux côtés des professionnels de santé, les pompiers, les préfectures, les agences régionales de santé et les collectivités ont joué un rôle déterminant et collectif. C'est cela, l'important. régionales de santé (ARS) des frais engendrés par la campagne de vaccination ont donné lieu à des discussions au tout début du printemps entre le Gouvernement et les représentants nationaux des collectivités territoriales.

En revanche, l'État intervient pour prendre à sa charge les frais supplémentaires engagés par les collectivités, tels que l'achat de matériel ou l'embauche d'agents supplémentaires dédiés. La compensation de ces éléments est intégralement assurée par les ARS dans le cadre des règles décidées avec les associations d'élus. Vous m'interrogez également sur l'avenir des centres de vaccination et je vous en remercie. Nous venons d'engager une campagne de rappel, elle concerne à ce jour les personnes âgées de plus de 65 ans et celles qui présentent des facteurs de risque, lorsque leur schéma vaccinal complet date de plus de six mois. La montée en puissance progressive de la campagne de vaccination initiale permet de gérer le volume des personnes concernées, en nous appuyant sur les professionnels de santé en ville. Les ARS ont commencé à ajuster le maillage des centres de vaccination, toujours en lien avec les élus locaux et les professionnels de santé-

n'est ni actée ni écartée à ce jour. En fonction de l'évolution des besoins, nous continuerons de faire appel aux collectivités qui le souhaitent et qui ont déjà répondu présentes, en connaissant les règles financières de leur mobilisation.

Sur le littoral, comme dans l'arrière-pays, en ville comme à la campagne, partout où je me rends, le problème est le même et il s'aggrave d'année en année : nous manquons de professionnels de santé, en particulier de médecins, et d'équipements. La désertification médicale prospère ! Dans ce contexte, les élus locaux déploient des efforts considérables pour assurer une couverture médicale minimale à nos concitoyens : ils construisent des maisons de santé, ils recrutent des médecins, ils financent même parfois certains équipements, comme l'hélicoptère du SAMU. Ils persistent à réclamer des moyens, souvent je pense par exemple au scanner de la ville de Limoux. Alors que la population augmente sur l'ensemble du département et que les personnes vivent plus longtemps, les moyens et les services diminuent. Faute d'offre médicale suffisante en soins de ville comme en soins hospitaliers, la patientèle fuit inévitablement vers les métropoles montpelliéraine et toulousaine,

Bien qu'ils aient confiance en leurs élus locaux, ces derniers ne peuvent pas tout régler seuls et, surtout, ils ne peuvent pas se substituer en permanence à l'État. La problématique médicale devient un enjeu majeur de développement et d'aménagement du territoire.

Monsieur le sénateur Sebastien Pla, le défi démographique que nous avons à relever aujourd'hui est grand : le nombre de médecins est en baisse régulière depuis 2010 et cette baisse est susceptible de se poursuivre jusqu'en 2025 dans de trop nombreuses

pour améliorer l'accès aux soins, en particulier dans les territoires qui en ont le plus besoin. Le déploiement de l'exercice coordonné représente par exemple un fort levier d'attractivité. À plus courte échéance, pour libérer du temps médical et redynamiser les soins de proximité, nous créons 4 000 postes d'assistants médicaux pour seconder appuyer les médecins dans un ensemble de tâches administratives et nous facilitons le déploiement de 400 médecins généralistes dans des territoires prioritaires. La dynamique autour des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) apporte également une réponse structurelle et rapide pour faire face aux besoins locaux de santé. Dans votre région, (ARS) travaille en concertation avec l'ensemble des acteurs et des élus pour garantir la pérennité d'une offre de soins de proximité. À Tuchan, l'action combinée des médecins de la CPTS et de l'ARS a conforté la maison de santé pluridisciplinaire, en intégrant deux médecins généralistes supplémentaires pour un bassin de vie de 2 000 habitants. À Narbonne, une grande concertation a permis de créer la CPTS du Grand Narbonne, qui a été mobilisée, je le précise, comme vaccinodrome, ainsi que deux maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers prioritaires de la

Madame la ministre, je pense que c'est sans surprise que vous avez pris connaissance de l'objet de ma question. Nous sortons d'un épisode électoral qui a suscité bien du mécontentement, tant de la part des électeurs que des maires en charge de l'organisation de ces élections.

Les maires n'ont cessé de relayer ce manquement à la citoyenneté. Malgré une société numérique, il faut savoir que nombre de Français attachent une grande importance à la réception et à la lecture des bulletins de vote et des professions de foi. Il est légitime de penser que les déboires de cette distribution ont pu conforter nos concitoyens dans leur décision de rester chez eux. Cela a pu contribuer au désintérêt général

Plutôt que de nous affliger un peu plus encore de ce constat, je souhaite à l'occasion de cette question faire une proposition. Est-il envisageable- et envisagé -de départementaliser cette mission, en confiant aux préfets de département l'organisation de la mise sous pli et de la distribution, en s'appuyant de nouveau sur les communes chefs-lieux de canton pour gagner en proximité et en qualité ? À la veille des grands rendez-vous électoraux de 2022, il me semble qu'il est temps d'agir.

ne peut exclusivement être la conséquence des dysfonctionnements- intolérables, je vous rejoins -dans l'acheminement de la propagande. Dans la Drôme, ces dysfonctionnements ont été le résultat d'une double défaillance celle du routeur KOBA et celle du distributeur Adrexo. KOBA n'a pas réussi à mettre sous pli dans les délais la totalité des documents de propagande pour le second tour, mettant en difficulté la société Adrexo son côté, n'est pas parvenue à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour rattraper ce retard. Afin que de tels incidents ne se reproduisent pas, le ministre de l'intérieur a pris deux décisions. D'une part, les différents lots qui liaient le ministère de l'intérieur à la société Adrexo ont été résiliés le 13 août dernier. Jusqu'au 31 décembre 2021, un marché passé en urgence impérieuse avec La Poste permettra le bon acheminement de la propagande- je pense aux élections partielles. Ensuite, un nouveau marché pérenne sera passé selon la procédure de droit commun. Cet accord-cadre tiendra compte des principales conclusions formulées par la commission des lois du Sénat dans son rapport paru le 21 juillet dernier. D'autre part, le ministère de l'intérieur a décidé que la mise sous pli de la propagande électorale serait, sauf exception dûment justifiée, réinternalisée sous la responsabilité directe des préfectures de département. Autrement dit, deux modalités de mise sous pli sont dorénavant acceptées : la mise sous pli réalisée en régie préfectorale et celle qui est déléguée par les préfectures à des communes volontaires une convention. Ces décisions me semblent être de nature à sécuriser le mieux possible les opérations relatives à l'acheminement de la propagande électorale, élément essentiel à l'exercice par chacun du droit de vote. La parole

sur les deux millions de nos concitoyens qui reçoivent chaque année des courriers, des mails et des SMS frauduleux les incitant à communiquer leurs données personnelles et bancaires, 300 000 en sont malheureusement victimes. Ces Ces techniques dites d'hameçonnage ou, en anglais, de consistent, pour le fraudeur, à se faire passer pour un organisme familier- banque, administration fiscale, caisse de sécurité sociale -afin de tromper le destinataire. La crise sanitaire a représenté une opportunité majeure pour ce type de criminalité, les fraudeurs ayant profité de l'intensification des usages numériques pour démultiplier leurs attaques, notamment pendant les phases de confinement.

Certaines bases de données en ligne vont même jusqu'à proposer à la vente des millions d'adresses de messagerie et de numéros de téléphone pour quelques centaines d'euros. Des méthodes prêtes à l'emploi sont disponibles en ligne et permettent de professionnaliser les attaques, en les rendant toujours plus difficiles à détecter pour les victimes. L'hameçonnage, quel que soit son type, est aujourd'hui l'une des formes les plus virulentes de fraudes et d'attaques informatiques. Madame la ministre, quels moyens sont mis en place pour mieux informer et protéger nos concitoyens et surtout pour mieux lutter contre ce type de fraude ?

Les forces de sécurité intérieures sont mobilisées contre les nouvelles menaces qui en découlent- vous les avez parfaitement résumées. Le Gouvernement a mis en place un réseau d'enquêteurs spécialisés comprenant plus de 2 900 enquêteurs formés aux investigations sur internet et les réseaux sociaux, plus de 700 primo-intervenants en cybercriminalité et plus de 460 investigateurs en cybercriminalité. Nous poursuivons aussi l'adaptation du dispositif de lutte contre les cybermenaces avec la création du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace qui regroupe les unités spécialisées intervenant sur ces thématiques et du réseau Cybergend constitué de plus de 10 000 enquêteurs formés aux cybermenaces. J'adresse mon soutien aux agents de la direction centrale de la police judiciaire qui, en mai 2021, en lien avec les douanes et la police aux frontières, ont porté un coup d'arrêt aux activités du forum Le Monde Parallèle, après avoir réussi à démanteler les plateformes illicites du francophone La Main Noire en juin 2018 et

signalements d'escroqueries au premier semestre 2021. Le numéro Info Escroqueries, qui est chargé d'informer et d'orienter les personnes victimes d'une escroquerie, a traité 25 786 appels

renforcer le traitement judiciaire des escroqueries en ligne et de démanteler les organisations criminelles. Enfin, le Gouvernement a lancé, dès 2017, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr pour guider et accompagner les victimes. Je les invite à la consulter autant que de besoin. La parole

La volonté affichée par le Gouvernement d'assurer l'égalité de chaque citoyen devant le droit à la sécurité impose une juste adéquation des moyens aux besoins de sécurité de la population, ce qui nécessite notamment l'affectation en nombre suffisant de militaires ou de ressources pour la réserve opérationnelle. de la création de 40 postes en quatre ans, mesure qui est unanimement saluée dans ce département où la croissance démographique est très vive sous la double influence de Lyon et de Genève, force est de constater qu'une cinquantaine de postes ne sont pas pourvus à ce jour. À ce constat s'ajoute l'épuisement, depuis le 1septembre, des ressources budgétaires de la réserve opérationnelle, qui empêche toute action de renfort, par exemple lors des manifestations sportives ou culturelles. Auvergne-Rhône-Alpes pourrait prochainement bénéficier de l'affectation d'environ 70 militaires en sortie d'école, leur répartition dans chacun des départements de la région ne permettra pas- vous en conviendrez -de pourvoir les 50 postes vacants dans l'Ain. Investis de la mission de sécurité et de paix publiques, les militaires peinent aujourd'hui à l'exercer dans des conditions satisfaisantes dans chacun des domaines qui relèvent de leur compétence. De nombreuses opérations de sécurité sont en effet touchées par cette situation, à l'instar des opérations de sécurité routière destinées aux plus jeunes. C'est pourquoi, dans un souci de maintien de l'ordre républicain, de protection de la population et de sécurité des territoires aindinois, je souhaite que vous me renseigniez sur les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour remédier à cette situation inquiétante et permettre aux unités de gendarmerie de l'Ain de bénéficier des effectifs adaptés aux réalités locales, dans l'attente de l'affectation des militaires issus des écoles. La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur

qui prévoyait la création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires d'ici à 2022. Dans le département de l'Ain, les effectifs affectés en brigades territoriales ont ainsi augmenté plus rapidement que la population. En effet, entre 2017 et 2020, la population a augmenté de 2,7 contre 4,7 % pour le nombre de gendarmes chargés d'assurer sa protection, soit 41 équivalents temps plein supplémentaires. Le taux de criminalité a d'ailleurs diminué de 19 % alors que le taux d'élucidation d'affaires a augmenté de 12 % sur la même période. Vous le savez, monsieur le sénateur, le Gouvernement s'engage et continuera de s'engager de façon importante en matière d'effectifs dans votre département. Vous mentionnez également des tensions sur l'emploi de la réserve opérationnelle. Elle a en effet connu une activité plus dense, en particulier à la suite de l'attentat de Nice du 29 octobre 2020. L'apport de cette entité dans l'offre globale de sécurité est fondamental. Ainsi, le 14 septembre, le Président de la République a annoncé, lors de la clôture des travaux du Beauvau de la sécurité, une augmentation substantielle et historique du nombre de réservistes opérationnels de la gendarmerie, appelé à être porté à 50 000 dans les toutes prochaines années. Ce sont autant de femmes et d'hommes qui pourront s'engager au service de nos concitoyens pour toujours plus de tranquillité et de sérénité au coeur de chaque territoire. La parole

qui vise à mieux accompagner l'investissement dans ces établissements. Aujourd'hui, près de 130 projets de modernisation sont déjà inclus dans ce plan, mais il est malheureusement trop restrictif pour les abattoirs nouveaux ou en réouverture, comme celui de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Fermé depuis 2011 à la suite du départ de l'entreprise Bigard, cet abattoir devrait rouvrir d'ici à la fin de l'année 2021. Situé au milieu du pays de Bray, au carrefour de nombreuses activités rurales, il collaborera avec les éleveurs de proximité.

Cette mise à disposition tarde à se mettre en place et compromet la réouverture prévue avant la fin de l'année. Monsieur le ministre, comptez-vous intégrer l'abattoir de Forges-les-Eaux dans le plan Abattoirs ? Cela permettrait d'alléger le coût de cette réouverture.

sans difficulté majeure, ce qui permet d'envisager l'attribution d'un agrément conditionnel d'ici à la fin de l'année 2021, si les travaux sont réalisés selon le calendrier présenté.

et que la pandémie de covid a conforté une agriculture de proximité et durable, il nous paraît nécessaire que cette agriculture puisse être défendue à l'échelon européen avec la même cohérence. Les négociations de la future politique agricole commune (PAC) pour 2023-2030 se terminent dans tous les États membres. Le plan stratégique national agricole doit être envoyé à la Commission européenne avant le 1 janvier 2022, avec effet au 1 janvier 2023- autant dire demain Dans ce contexte, l'agriculture de montagne et son élevage sont très caractéristiques du modèle agricole français durable, ancré dans les territoires et avec une forte valeur ajoutée environnementale, mais ils sont aussi plus fragiles et dépendants des mesures européennes de soutien. Or ce modèle de l'agriculture de montagne suppose, plus que jamais, un engagement majeur et diversifié des politiques publiques européennes en faveur de l'agriculture, de l'environnement et de la ruralité. Plus concrètement, la qualité de l'agriculture de montagne perdure grâce au maintien des aides couplées, de l'éligibilité des surfaces agropastorales aux aides surfaciques, de l'aide aux jeunes agriculteurs et des aides destinées à la modernisation des bâtiments. De la même manière, l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) mériterait d'être renforcée et ciblée davantage sur l'élevage. Il s'agit en effet de rémunérer à leur juste valeur les services environnementaux rendus par des exploitations herbagères et des surfaces pastorales. compte tenu des risques climatiques accrus et du fait que les orientations de la PAC sont prévues pour durer jusqu'en 2030, l'agriculture de montagne requiert la mise en place de modes de gestion des risques climatiques mutualisés et performants afin que nous puissions continuer de proposer un modèle durable et d'attirer les jeunes éleveurs. Aussi, monsieur le ministre, ma question est la suivante quelles mesures concrètes allez-vous proposer dans le plan stratégique national pour continuer de faire vivre, par des mesures de soutien, l'agriculture et l'élevage de montagne ? La parole